séance est reprise. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, M. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains, a demandé le retrait de l'ordre du jour du jeudi 23 février 2017 de la proposition de loi permettant un exercice territorialisé de compétences au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cinquante communes au moins. Acte est donné de cette demande. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables

L'Assemblée nationale a confirmé hier son vote, en nouvelle lecture. Me voici donc aujourd'hui, une nouvelle fois, devant vous à l'occasion de l'examen de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi de ratification des trois ordonnances qui permettront à la collectivité de Corse de voir le jour,

même si, je ne vous le cache pas, mon espoir s'amenuise, vous convaincre d'adopter ce projet de loi, qui est, soyez-en convaincus, un bon texte, utile et même nécessaire pour la Corse et les Corses. Je souhaite, en préambule, vous rappeler que les ordonnances soumises à votre ratification ne font que permettre la mise en oeuvre de la future collectivité

vous rappelle en outre que les élus de l'Assemblée de Corse ont appelé de leurs voeux à une très forte majorité ... À 80 % ! ... et toutes tendances politiques confondues, le 12 décembre 2014, à la création de cette collectivité unique. Ces ordonnances complètent et précisent les règles budgétaires, financières et comptables applicables à la collectivité de Corse- c'est l'objet de l'ordonnance n° 2016-1561 les mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse, au travers de l'ordonnance n° 2016-1562, et les diverses mesures électorales applicables en Corse, avec l'ordonnance n° 2016-1563.

et députés souhaitaient l'adoption lors du débat relatif à la loi NOTRe. Je veux également indiquer que les amendements de votre commission des lois, qui apportaient des précisions rédactionnelles intéressantes, ont été repris par l'Assemblée nationale. À ce titre, je ne citerai que les deux améliorations les plus fondamentales que l'on doit aux parlementaires.

de mieux coordonner l'action publique et la solidarité financière entre la collectivité de Corse, les communes et leurs intercommunalités. Ensuite,

Je me permettrai simplement de suggérer qu'une ultime assurance sur le sujet pourrait aussi leur être apportée aujourd'hui au Sénat, par la ratification des ordonnances.

J'entends souvent l'argument selon lequel il ne s'agirait pas de la collectivité souhaitée, voire rêvée. Je m'inscris en faux contre cet argument, qui n'est pas sérieux. L'article 30 de la loi NOTRe, qui institue la collectivité de Corse, n'est pas un article de principe. Il définit, en six pages de, dans le détail, sa substitution à la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Pour cela, il réécrit le chapitre du code général des collectivités territoriales relatif à la collectivité territoriale de Corse. Il n'est donc pas juste de prétendre que ce n'est pas la collectivité qu'il convenait de faire. Ces ordonnances ne sont que la déclinaison des principes votés dans le cadre de la loi ; elles se contentent, ainsi que je viens de le rappeler, de préciser ou d'adapter les règles. Ne pas accepter de les ratifier revient à dire que vous êtes opposés aujourd'hui à la création de ce que vous souhaitiez hier.

En ce qui me concerne, au nom du Gouvernement, je demeure fidèle à ce que j'ai toujours dit. Je n'entrerai pas dans les débats politiciens et j'accomplirai jusqu'à la fin de la législature- c'est bien la moindre des choses jusqu'à la fin de la législature- c'est bien la moindre des choses -le travail qui est le mien ; le fait qu'une quinzaine de jours nous séparent de la fin de cette législature n'entravera pas ma détermination. Le Gouvernement est au travail jusqu'au dernier

le 22 novembre 2016, afin qu'elles ne disparaissent pas de l'ordre juridique, ce qui empêcherait la création de la collectivité unique. Il est d'autant plus indispensable de les ratifier que les Corses attendent l'action du Gouvernement au service de leur territoire.

la gouvernance des institutions corses afin de la rendre plus efficace et d'améliorer, à moindre coût, les services publics. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, les raisons pour lesquelles je vous demande de nouveau et malgré l'échec de la commission mixte paritaire, d'adopter ce projet de loi de ratification. La collectivité unique de Corse doit voir le jour pour que les élus corses puissent mieux assurer l'avenir de l'île et de son peuple.

lorsque le gouvernement de l'époque- le ministre de l'intérieur s'appelait alors Nicolas Sarkozy -a proposé un texte qui créait une collectivité unique par fusion des départements.

Comme cela a été rappelé, le Gouvernement avait été habilité à prendre ces ordonnances par l'article 30 de la loi du 7 août 2015 Comme nos collègues députés, comme notre rapporteur et comme l'ensemble des groupes parlementaires, je constate que le Gouvernement a parfaitement respecté l'objet et les délais fixés par les ordonnances. Ces dernières respectent trois principes : assurer la neutralité budgétaire, comptable et financière de la réforme, pour permettre à la nouvelle collectivité de fonctionner au 1 janvier 2018

En fusionnant les deux conseils départementaux avec le conseil régional, ces trois ordonnances viennent parachever un processus entamé depuis près de vingt ans par le « processus de Matignon », engagé par En effet, la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse était restée au milieu du gué. En 2003, la fusion des collectivités avait été rejetée par les citoyens et citoyennes corses dans le cadre d'un référendum consultatif

qui ont été avalisés par une nouvelle délibération de l'Assemblée de Corse le 7 septembre 2016. C'est donc un processus de longue haleine, émanant des représentants de l'île et associant le Gouvernement et le Parlement,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons après l'échec de la commission mixte paritaire. Cet échec était prévisible, puisque le Sénat avait rejeté le projet de loi

Je partage le même optimisme que M. le ministre : j'espère que les opposants du 26 janvier auront changé d'avis. Nous allons profiter du présent débat pour finir de les convaincre. les convaincre. Je rappelle que le texte achève un processus de simplification des structures, tout en garantissant les spécificités corses. Il répond à une délibération de l'Assemblée de Corse prise en décembre 2014, qui appelait à la création de la collectivité unique.

les élus corses ont demandé à ce que l'on n'organise pas de consultation des électeurs corses : ils souhaitent que ce soit le Parlement qui mette en place la collectivité unique de Corse. Cela permet de répondre à l'argument des opposants, qui estiment qu'il est nécessaire d'organiser un référendum en Corse. En créant la collectivité unique, nous allons permettre à la Corse une évolution historique.

ans, va remplacer la région Corse et les deux départements corses. C'est en définitive l'aboutissement d'un très long processus, engagé par les statuts Defferre,

La fusion des différents échelons territoriaux s'inscrit pleinement dans le mouvement de décentralisation et de rationalisation de l'action publique, avec pour objectif de rapprocher la décision prise par les élus des populations locales. L'objectif est bien sûr économique- obtenir les meilleurs coûts -, mais il s'agit également de garantir une gouvernance plus solidaire et plus cohérente et de répondre efficacement aux attentes des habitants et aux déséquilibres des territoires.

je ne compte pas les divers syndicats et les nombreuses agences qui viennent ajouter à la complexité de l'architecture territoriale ! Je

paix sur l'île. J'ai bien entendu les arguments avancés par ceux qui s'opposent à cette évolution statutaire. Je comprends que le parti communiste reste sur une position très jacobine, mais

à l'Île-de-France, où l'on trouve des départements, des conseils de territoire, des communes, la région, la métropole ... Prenons exemple sur ce qui se passe en Corse pour simplifier notre organisation territoriale ! Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et républicain votera évidemment en faveur de ce projet de loi. La parole est à M.

26 janvier dernier. Par son insularité, par son histoire, la Corse dispose de spécificités, qu'il nous faut évidemment prendre en compte. Loin des images caricaturales que certains distillent, cette région est très loin d'être favorisée. Le revenu par habitant y est le plus faible du pays, et un Corse sur cinq vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. La question du coût de la vie est caractéristique des inégalités qui minent la Corse. Alors que l'on continue à consentir toujours plus de dérogations au grand patronat, avec, par exemple, 194 millions d'euros de réfaction de TVA accordée aux de la distribution sur l'île, les produits alimentaires y sont 9 % plus chers que sur le continent.

Le sous-investissement économique, au lieu de développer la filière maritime, a conduit l'État à liquider progressivement la SNCM, fleuron de l'économie corse. Le sous-investissement est aussi énergétique, avec 87 % de la consommation totale d'énergie issue d'approvisionnements extérieurs

entre les mains de quelques élus, est évidemment très préoccupant. En tout cas, ce n'est pas le signe d'une bonne santé démocratique ! Le danger d'un développement de l'affairisme, déjà malheureusement bien présent sur l'île, sera renforcé par ce recul du contrôle citoyen sur les élus. Nous n'acceptons pas ce glissement vers le modèle de l'Europe des régions, au détriment des nations. Cette mise en concurrence des territoires et des populations, poussée, on le sait, par les tenants de l'Europe fédérale, affaiblira la Corse et appauvrira ses habitants, qui, comme l'ont été les Grecs, seront dévorés par les directives bruxelloises. En fait, seuls les affairistes, les, oligarques confisquant les richesses de ceux qui, en Corse, travaillent dur, peuvent se réjouir d'un tel changement. Et ce n'est pas sans surprise que nous avons vu certains élus, jusque-là attachés au maintien de la Corse dans la République, céder aux sirènes des indépendantistes et des discours populistes. Enfin, je veux rappeler qu'un changement aussi profond de l'organisation territoriale de la Corse ne peut pas se décider dans le dos de la population. Une ratification par référendum après la tenue d'un grand débat public s'impose. En refusant obstinément cette consultation, vous exprimez une marque de défiance à l'égard des Corses, qui ne seraient pas jugés capables de donner leur avis sur leur avenir. Pour notre part, nous faisons pleinement confiance aux habitants et aux travailleurs de l'île et à leur capacité d'analyse. Ce dont ont besoin les Corses, c'est bien d'un renforcement de la solidarité républicaine, d'un nouveau plan de développement, alliant à la fois modernité, progrès social et réussites économiques, et non d'une énième réforme des institutions. Monsieur le ministre, il faut avoir le courage de la transparence ! Ce n'est pas en catimini, dans un hémicycle quasi désert, en fin de session parlementaire, qu'une telle décision peut être prise. Ouvrons largement le débat avec la population. Sortons des petits arrangements entre amis, sans avoir peur de la démocratie ! Pour l'heure, le groupe communiste confirmera son rejet de ces trois ordonnances.

nous y attendre, nous voici réunis pour une nouvelle lecture du projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la Corse. Mes chers collègues, il est nécessaire que ces ordonnances soient adoptées définitivement avant l'interruption des travaux parlementaires, pour permettre à la collectivité unique de Corse d'être installée rapidement, et ce dans les meilleures conditions. Le 12 décembre 2014, le principe d'une collectivité unique a été acté de manière républicaine et transparente par une très large majorité des élus de la Corse. Droite, gauche et nationalistes ont approuvé à 80 % la création de cette collectivité. Je tiens à rappeler que la création d'une collectivité unique a été sollicitée dès 2013 et 2014, à travers deux délibérations de l'Assemblée de Corse. le groupe du RDSE avait voté l'amendement relatif à la collectivité unique de Corse lors de l'examen de la loi NOTRe. C'est sur cette base que les ordonnances, qui doivent accompagner la mise en oeuvre de la collectivité unique au 1 janvier 2018, Très concrètement, il reste peu de temps pour construire un processus permettant à la future collectivité d'être opérationnelle au 1 janvier 2018. Les ordonnances permettent déjà d'avancer sur le plan de l'organisation administrative.

permettra de dégager des marges de manoeuvre pour améliorer la mobilité sur notre territoire, afin de lutter contre la désertification des territoires de l'intérieur et de montagne. Mes chers collègues, rien n'est figé. Une fois ces ordonnances ratifiées, le débat pourra être rouvert une loi spécifique à la Corse. nous pourrons notamment prévoir de construire une articulation spécifique entre les intercommunalités et la collectivité unique. Rien ne nous empêchera de corriger le tir et d'améliorer les procédures mises en place. La mise en place de la collectivité unique n'est désormais plus un sujet de débat. Elle est en passe de devenir une réalité et doit s'inscrire dans la durée. Aussi les ordonnances sont-elles une étape nécessaire dans la construction progressive d'un équilibre institutionnel et territorial qui permettra de relever de multiples défis pour les Corses et pour la Corse.

sans proposer un nouvel équilibre territorial. Le centralisme, au profit de la nouvelle collectivité et de ses représentants politiques, est réel. Ces ordonnances, qui découlent donc de la loi NOTRe, ne règlent pas les problèmes institutionnels, administratifs et financiers de la Corse. Monsieur le ministre,

Force est de constater aujourd'hui que ces ordonnances contraintes et étriquées ne nous permettent pas d'apporter les modifications nécessaires tant attendues en matière institutionnelle, électorale, financière et fiscale.

à savoir l'amendement relatif à la répartition du reliquat de l'enveloppe de la dotation de continuité territoriale qui a été introduit à l'Assemblée nationale

aux politiques publiques menées en faveur des territoires de montagne et de l'intérieur de l'île. Une étude consacrée à la remise à niveau de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires

vous me verrez, avec mes collègues du Sénat et de l'Assemblée nationale, continuer de défendre l'élaboration et l'adoption d'une loi spécifique à la Corse. La parole

À vos côtés, aux côtés des dirigeants de la collectivité de Corse, aux côtés des parlementaires corses, j'ai oeuvré pour la création de cette chambre qui permettra d'équilibrer le pouvoir entre Ajaccio et Bastia

Le scrutin est ouvert.

Merci